L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

faciliter le travail des acteurs de terrain qui exercent auprès des animaux, plutôt que de l'entraver ; refuser le credo « interdire et laisser mourir » et trouver, toujours, des solutions pour le bien-être des animaux et l'avenir des professionnels.

je regrette que la solution opérationnelle que nous avions proposée, à savoir l'élaboration d'une liste portant des interdictions progressives, ciblées et analysées espèce par espèce, après une consultation élargie, ait été refusée par les députés. montrer tous les animaux sauvages d'un coup posera de vraies difficultés : il sera compliqué de leur trouver des places d'accueil. Le Gouvernement ne le réalise qu'aujourd'hui : c'est un peu tard Toutefois, le Sénat a obtenu un délai de transition de sept ans, pour laisser le temps aux professionnels de s'organiser. Aucune interdiction de détention d'un animal ne sera prononcée sans la proposition, pour les animaux, d'une solution d'accueil qui garantisse leur bien-être. À défaut, des dérogations seront mises en oeuvre. C'est la moindre des attentions que nous devions aux circassiens, que nous respectons et qui crient leur désespoir. leur doit est piétiné lorsque certains animalistes les traitent de « maltraitants » et s'opposent physiquement à l'exercice de leur activité pourtant légale, encadrée et contrôlée. Un véritable délit d'entrave doit être instauré pour faire cesser cette guérilla dangereuse et inacceptable. Le Sénat a déjà voté une proposition de loi dans ce sens ; la balle est dans le camp des députés. Je veux insister sur un point : les voleries ne relèvent pas de cette interdiction dès lors qu'elles ne sont pas considérées comme itinérantes, mais mobiles. Cela a été réaffirmé en commission mixte paritaire concerne les parcs zoologiques aquatiques, auxquels le législateur est très attaché, le texte garantit que les vingt et un dauphins et les quatre orques présents en France pourront être conservés dans ces établissements si ceux-ci s'engagent dans des programmes scientifiques reconnus ; ils pourront présenter le contenu et les résultats de leur recherche au public. Cela évitera que ces cétacés finissent dans des piscines de luxe à l'autre bout du monde ou qu'ils soient euthanasiés. C'était, là encore, une ligne rouge pour le Sénat, qui a tenu bon. Sur les animaux de compagnie, la lutte contre l'abandon a été érigée en priorité, avec la mise en place d'un certificat d'engagement signé par l'acquéreur, en lien avec un délai de réflexion de sept jours avant l'achat, dans des conditions précisées par décret de manière à ne pas créer de difficultés pour la tenue de certains événements, comme les foires. Je pense aussi aux nouvelles sanctions et aux moyens renforcés alloués à la lutte contre les trafics. Un encadrement strict des offres de cession en ligne d'animaux de compagnie est acquis : le contenu des annonces sera vérifié et labellisé par ces plateformes, qui en seront responsables. Ce point est une avancée historique, que l'on S'agissant des animaleries, notre assemblée a rétabli la vente de tous les animaux de compagnie, à l'exception des chiots et des chatons ; des dérogations seront accordées aux refuges, qui pourront proposer à l'adoption leurs animaux en magasin. Nos arguments ont convaincu

Je me félicite de la reconnaissance législative des associations sans refuge, alors que leur existence même était menacée au sortir de l'Assemblée nationale. Ces bénévoles sont des acteurs de terrain essentiels. Je me réjouis enfin des mesures renforcées que nous avons proposées contre la zoophilie et la zoopornographie, ainsi que de l'abandon de l'idée absurde d'obliger les maires à faire stériliser les chats errants sans compensation financière ou d'imposer la construction d'une fourrière dans chaque commune, autre ligne rouge pour le Sénat. Tous ces apports sénatoriaux aboutissent à un texte équilibré et opérationnel, plus pragmatique et moins idéologique, qui me semble répondre aux objectifs partagés par le plus grand nombre pour améliorer la condition animale. Pour ma part, je n'exprimerai qu'un seul remerciement, celui de m'avoir placée sur le chemin de professionnels exceptionnels, passionnés et passionnants, qui oeuvrent pour le bien-être et la connaissance des animaux, ainsi que le rapprochement de ceux-ci avec l'homme. Je vous invite, mes chers

je sais leur attachement à ces animaux, nous sommes tous conscients que cette évolution peut être douloureuse et nous serons à l'évidence pleinement à leurs côtés pour que cette transition soit la plus sereine possible.

bien sûr, mais aussi pour certains programmes scientifiques qui devront être validés par le Gouvernement. Nous serons évidemment d'une grande vigilance sur les programmes que nous autoriserons et sur leur évaluation.

pour que chacun soit pleinement conscient de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis d'un animal de compagnie. C'est pourquoi je me félicite de la création, par ce texte, d'un certificat d'engagement et de connaissance pour toute acquisition d'un animal de compagnie ou d'un équidé. Le Gouvernement aura à coeur de publier les textes d'application nécessaires à sa mise en oeuvre dans les plus brefs délais.

C'est une avancée majeure pour nos animaux de compagnie. Toujours dans cette optique, vous avez acté l'encadrement de la vente en animalerie à partir de 2024. Cela nous permettra de lutter contre les achats impulsifs de chiots et de chatons et de limiter ainsi les risques d'abandon. Il faut toujours rappeler que l'objectif de ces mesures est bien d'opérer une prise de conscience collective et de l'accompagner. Détenir un animal de compagnie, c'est une joie qui concerne un foyer sur deux en France- nous avons là un important levier de médiation et de participation à cette réflexion

Pour toucher un public plus large, ce texte prévoit qu'une sensibilisation à l'éthique animale sera dispensée lors du service national universel, mais aussi dans le cadre de l'enseignement moral et civique, à l'école primaire, au collège et au lycée.

Pour simplifier l'action des communes dans la mise en oeuvre de cette politique publique, vous avez actualisé le dispositif des fourrières et de la gestion de l'errance animale. C'était également une attente extrêmement forte.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire,

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires avait quelques points de divergences avec le texte issu du Sénat, car celui-ci remettait en question des avancées nous mettant pourtant tout juste au niveau de pays plus protecteurs en Europe. Cependant, nous avions salué certains apports de notre commission, notamment sur la question des sanctions ou sur le statut donné aux associations sans refuge. Quant à cette ultime version du texte, nous regrettons toujours qu'elle ne traite pas de sujets essentiels pour la lutte contre la maltraitance, comme ceux de la faune sauvage victime

très attendue par les associations, avec une exception bienvenue pour les animaux issus des refuges, dans le cadre d'un partenariat entre animaleries et associations, afin de favoriser les adoptions de chats et chiens abandonnés. Ce compromis nous paraît plutôt pertinent. L'introduction d'un délai de réflexion de sept jours avant l'achat d'un animal de compagnie et le certificat d'engagement et de connaissance pour les futurs détenteurs d'animaux sont des mesures utiles, qui permettront une évolution bienvenue des pratiques pour prévenir la maltraitance animale. Concernant le renforcement des sanctions, nous nous félicitons que les sévices et les atteintes sexuelles soient plus lourdement punis. De nouvelles circonstances aggravantes ont été créées afin de mieux protéger les animaux ainsi que les enfants, lorsque ces actes sont malheureusement perpétrés sous leurs yeux. Enfin, nous ne pouvons que nous réjouir du rétablissement par les députés de l'interdiction de l'acquisition de mammifères marins et de leur reproduction dans les delphinariums, dans un délai de cinq ans, et de l'interdiction de la détention d'animaux sauvages par les cirques itinérants, dans nous souhaitions aller plus loin et prohiber la présence d'animaux sauvages dans l'ensemble des spectacles, fixes ou itinérants, et ce dans des délais plus brefs, mais il s'agit déjà d'une avancée majeure, qu'il faut reconnaître. Nous appelons tout de même à la vigilance quant au risque de sédentarisation des cirques itinérants : les cirques fixes n'étant quant à eux soumis à aucune interdiction, ils pourront toujours posséder des animaux sauvages. À l'État maintenant de faciliter cette transition et d'accompagner les cirques et les établissements animaliers vers des spectacles sans animaux. Enfin, nous nous réjouissons de l'interdiction de l'élevage de visons et d'animaux d'espèces non domestiques destinés à l'industrie de la fourrure, avec effet immédiat dès la promulgation de la loi.

inscrite dans le texte initial, pour les maires et les intercommunalités de prendre en charge ce problème, il nous paraissait légitime que l'État, en parallèle, engage des moyens supplémentaires pour soutenir les collectivités dans cet objectif de politique publique. Sur cette question, il faut aller vite. Nous suivrons de près les travaux de l'Observatoire de la protection des animaux de compagnie, dont nous espérons qu'il alimentera judicieusement le rapport prévu à l'article 3, lequel devra prévoir des propositions de financements pérennes pour la mise en place de ces campagnes de stérilisation. Bien sûr, beaucoup reste à faire, notamment sur un autre aspect fondamental de la souffrance animale : l'élevage industriel. Nous en sommes convaincus, lutter contre la souffrance animale passe par un changement de notre modèle agricole et en particulier Nous y reviendrons dans d'autres débats, je n'en doute pas. Pour conclure, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera pour ce texte, certes encore timide sur certains sujets, mais qui acte des progrès majeurs pour mieux protéger les animaux de la violence et de l'abandon. Je vous remercie,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, malgré ses imperfections et ses manques, cette proposition de loi constituait une avancée pour la lutte contre la maltraitance animale, car sur ce sujet nous partons de très loin.

D'abord, les spectacles avec des animaux sauvages seront finalement interdits dans les delphinariums en 2026, malgré des dérogations, et dans les cirques itinérants en 2028. À ce sujet, je tiens à souligner la proposition de Mme la rapporteure, acceptée en commission mixte paritaire, de trouver d'ici à 2028 une solution pour accueillir ces animaux de cirque au lieu de les euthanasier comme le prévoyait l'Assemblée nationale. Il en va de même pour la fin de la vente de chats et de chiens en animalerie à partir de janvier 2024. Nous sommes plus partagés sur cette question, car nous avons conscience que cela peut accroître le risque d'augmentation du nombre d'élevages clandestins ; il est impératif de renforcer les contrôles. Cela étant, on sait que les animaux vendus en animaleries sont issus souvent d'élevages d'Europe de l'Est, où ils sont détenus dans des conditions déplorables, sevrés trop tôt, ce qui entraîne des conséquences comportementales, et transportés dans de très mauvaises conditions ; d'ailleurs, beaucoup meurent au cours du trajet. proposition de loi s'est cantonnée aux mesures les plus consensuelles et certains sujets n'ont pas été abordés, mais il est important qu'un texte soit voté pour apporter un début de réponse aux attentes de nos concitoyens. En effet, il n'est plus acceptable que les animaux soient considérés comme des objets ou de simples marchandises dont on fait la promotion, que l'on offre sans réfléchir aux conséquences et que l'on peut jeter après un achat compulsif ou non raisonné. Il n'est plus acceptable que des animaux sauvages soient tenus en captivité et exhibés dans un cadre et un environnement qui ne sont pas les leurs. Dans le même temps, il nous faudra être vigilants afin que certaines pratiques ne perdurent pas du fait des lacunes que ce texte laisse subsister ; encore une fois, la parole du politique en sortirait grandement affaiblie.

Au-delà du texte en lui-même, je pense que cet accord en commission mixte paritaire nous oblige. Il nous oblige à une réflexion et à une action plus globale en faveur des animaux. Il nous oblige aussi à débattre de sujets qui crispent et à faire évoluer certaines pratiques. Je pense à la nécessité de revoir complètement notre modèle d'élevage intensif et notre rapport aux animaux que l'on dit « de rente », avec les agricultrices et les agriculteurs, mais je pense aussi à la protection d'espèces en voie de disparition et à la fin de l'usage irraisonné des pesticides dont l'impact sur la biodiversité est dévastateur. Rappelons que la biodiversité est une condition indispensable de la vie sur Terre. je l'ai dit en première lecture, je ne suis pas favorable à la politique des petits pas ; pour autant, je pense sincèrement que la cause animale est un sujet que nous ne pourrons plus occulter et qu'il est urgent d'en débattre ici, car il s'agit d'une question éminemment politique. Ne nous y trompons pas, la société capitaliste, qui se traduit par l'exploitation de l'homme et de l'environnement, porte aussi préjudice aux animaux. La recherche effrénée du profit se fait au détriment de la vie humaine,

Nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à attendre que nous nous saisissions véritablement de la question de la maltraitance animale. Il nous faut maintenant aller plus loin.

Nous voterons cette proposition de loi, en espérant qu'elle ne sera qu'une première étape à la fois dans la lutte contre la maltraitance animale et dans une réflexion sur notre rapport

Entre les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, un dialogue apaisé et des échanges fructueux ont eu lieu. Nous pouvons d'autant plus nous en féliciter que le sujet traité, particulièrement délicat, est souvent à l'origine de débats passionnés.

Les relations entre l'homme et l'animal ont connu au cours du temps des évolutions considérables dans notre pays. Autrefois, la force des animaux était la principale énergie disponible, en particulier pour l'agriculture et les transports. L'exploitation des énergies fossiles, puis renouvelables, les a libérés de cette servitude, mais ces relations se perpétuent de multiples manières, principalement dans l'élevage, qui a lui aussi connu de profonds changements, et pour l'agrément des humains.

d'abord par la société, puis par le législateur dans la loi du 10 juillet 1976. Par voie de conséquence, la protection du bien-être animal a été continuellement renforcée au fil des années par la loi et le règlement.

Au vu de l'évolution des mentalités, eu égard aux souffrances provoquées par le dressage et le travail de ces animaux, ainsi que par leur vie itinérante, il était nécessaire Toutefois, et le Sénat y fut attentif, il fallait procéder de manière ordonnée et laisser suffisamment de temps aux professionnels pour s'adapter à cette interdiction et pour trouver des hébergements convenables aux animaux. Le texte que nous votons aujourd'hui comporte des délais appropriés. L'instauration de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, composée d'experts, ajout du Sénat, figure également dans le texte final. deuxième point concerne la vente d'animaux de compagnie. À côté de la vente en animalerie s'est développée, grâce à internet, la vente en ligne entre particuliers. Le texte voté par les députés interdisait la vente en animalerie d'ici à 2024 afin de favoriser l'adoption des animaux de refuges. Cette position, à laquelle les députés se sont montrés fermement attachés en commission mixte paritaire, est assez discutable, eu égard au fait que la vente en animalerie est déjà soumise à une réglementation rigoureuse, comme nous avions eu l'occasion de le dire ici. Il est à craindre que la vente en ligne de particulier à particulier sur des plateformes comme Le Bon Coin, qui sont beaucoup moins réglementées, ne bénéficie de cette interdiction. Nous pouvons en revanche nous satisfaire du maintien de l'amendement sénatorial visant à interdire la présentation d'animaux dans les vitrines des animaleries.

Dans l'ensemble, ce texte améliore de façon concrète la situation des animaux dans notre pays. Il était en effet nécessaire d'adapter la législation aux évolutions de la société et de répondre ainsi à une attente de nos concitoyens. J'espère que son adoption pourra contribuer à l'apaisement dans ce domaine où, je l'ai dit, les oppositions peuvent être virulentes et parfois donner lieu à des débordements. Pour conclure, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, une majorité du groupe Union Centriste votera cette proposition de loi.

On oublie trop souvent le travail de concertation menée par députés et sénateurs, qui parviennent à s'entendre sur des textes communs au-delà des divergences politiques et de l'agenda électoral. Aujourd'hui, nous renforçons la protection des animaux ; nous pouvons nous réjouir de ce travail commun et fructueux. Certaines dispositions vont, je le pense, dans le sens de l'Histoire. Elles permettront de rattraper en partie le retard accumulé par la France dans ce domaine, retard qui nécessitait une mise à niveau rapide et ambitieuse. Les mentalités ont évolué et il est sain que notre législation s'y conforme. Ainsi, il sera interdit, dans un délai de deux ans, d'acquérir, de commercialiser ou de faire se reproduire des ours et des loups dans des spectacles itinérants et tout animal non domestique en vue de la présentation au public. Dans un délai de cinq ans, l'interdiction de la détention, de la reproduction en captivité et, bien sûr, des spectacles de cétacés entrera en vigueur. Dans un délai de sept ans, il sera interdit de détenir, de transporter ou de produire des spectacles incluant des animaux non domestiques dans les cirques itinérants. ailleurs, la promulgation de la loi marquera la fin de l'élevage des visons d'Amérique et de tous les animaux non domestiques élevés pour leur fourrure. Enfin, une liste révisée tous les trois ans déterminera les espèces d'animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie.

plus de 100 000 chaque année. En la matière, la palme du record européen nous fait honte et nous oblige à agir sans attendre. Toute première acquisition d'un animal de compagnie sera donc désormais soumise à la signature d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce à un délai minimal de sept jours de réflexion. Il ne sera plus possible ni de vendre ni de donner un animal de compagnie à un mineur sans le consentement préalable de ses représentants légaux. Les apports du Sénat ont été conservés sur ces deux points pour mieux décourager les achats impulsifs, qui sont souvent la cause des abandons. Dans le même objectif, comme mon groupe le défendait, les chiens et les chats ne pourront plus être vendus en animalerie à compter de 2024. Des chiens et chats abandonnés, destinés à l'adoption, pourront toutefois être présentés en animalerie par les bénévoles d'associations de protection des animaux. Pour les autres animaux, la vente restera autorisée, mais non la présentation en vitrine extérieure. La vente en ligne d'animaux de compagnie sera mieux encadrée, de même que les informations figurant sur l'offre de cession. Nous nous félicitons d'ailleurs du maintien dans le texte final de notre amendement visant à introduire dans l'annonce le nombre de portées de la femelle au cours de l'année écoulée. Ces mesures envoient un message clair : il faudra désormais faire appel à des associations ou à des éleveurs respectueux du bien-être animal, en mesure d'accompagner chaque nouvel acquéreur. Les animaux ne sont pas des biens de consommation courante ; ils doivent être considérés à chaque étape de leur vie comme des êtres doués de sensibilité. Enfin, l'arsenal juridique a été renforcé pour mieux lutter contre la maltraitance animale. La levée du secret professionnel du vétérinaire permettra de porter à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à des actes de cruauté ou à de mauvais traitements envers un animal. Les peines ont été aggravées dans les cas d'atteintes sexuelles, d'abandon avec mise en danger de la vie de l'animal, de mise à mort d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, de même que dans les cas de sévices graves ou d'actes de cruauté.

Malheureusement, il est souvent difficile de prouver l'élément intentionnel. C'est pourquoi le renforcement des dispositions pénales devait s'accompagner de mesures de prévention susceptibles de faire durablement évoluer les mentalités. Le stage de prévention et de lutte contre la maltraitance animale viendra remplacer ou compléter les peines d'emprisonnement, l'objectif étant de réduire les récidives grâce à une plus grande sensibilisation. En matière de prévention, on n'en fait jamais trop : nous sommes donc satisfaits de constater qu'un module consacré à l'éthique animale figurera au programme du service national universel et de celui de l'enseignement moral et civique dans le primaire et le secondaire. Aussi, vous l'aurez compris, le groupe du RDSE votera sans réserve cette proposition de loi. S'il lui a été reproché de ne pas balayer tous les sujets relatifs au bien-être animal, elle est le fruit d'un travail de concertation transpartisan et porte en elle des avancées qu'il nous est impossible de renier. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les résultats des travaux du Sénat sur ce texte à l'issue de sa première lecture étaient, à divers égards, décevants. de la commission mixte paritaire redonnent de la consistance à cette proposition de loi, mon engagement envers le bien-être animal m'oblige à y relever certaines lacunes. L'interdiction de l'exploitation des animaux non domestiques à des fins de divertissement constitue une avancée dans notre relation avec les animaux. Je regrette cependant la longueur des délais accordés aux acteurs concernés pour mettre fin à certaines pratiques. Bien que la reconversion nécessite du temps, la possibilité d'acquérir et de faire reproduire des animaux pendant encore deux ans est injustifiable. Que deviendront-ils dans cinq ans, une fois l'interdiction devenue effective ? Je tiens toutefois à féliciter les cirques ayant déjà mis en place des alternatives innovantes à cette exploitation. Je pense, entre autres, à l'introduction dans leurs spectacles d'hologrammes animaliers. Se divertir sans causer de souffrance, c'est possible, et les cirques le prouvent.

constituent des avancées louables. L'offre immense que constitue ce marché favorise les acquisitions non réfléchies et donc les abandons, au nombre de 300 000 par an. Cependant, ces progrès ne doivent pas nous faire oublier le bilan insuffisant du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le sujet. des mesures relatives à la lutte contre la maltraitance des animaux d'élevage ? Les propositions de vidéosurveillance des abattoirs, d'encadrement du transport et d'amélioration des conditions de vie sont absentes du texte. Le constat est identique pour la faune sauvage. République, à des fins électorales évidentes, offre des avantages exagérés aux chasseurs, au détriment des animaux, de la nature et de notre sécurité. En instaurant une différenciation entre les animaux qu'il n'est plus possible de maltraiter et les autres, ce texte n'atteint hélas que partiellement son objectif. Une réforme globale et ambitieuse du droit animal serait la bienvenue. Je voterai toutefois pour ce texte. Oui,

Durant les semaines d'examen du texte dans les deux chambres, jusqu'à la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire aujourd'hui au Sénat, nous avons tous constaté la mobilisation, l'engagement et l'émoi que pouvait susciter la maltraitance animale. Comme sur la majorité des sujets sociétaux, les oppositions ont été fortes et les débats ont été animés dans l'hémicycle et lors des travaux de préparation de la commission mixte paritaire. La vitalité de notre démocratie passe aussi par ces échanges et ces réflexions sur la place et les droits des animaux. L'aboutissement de ce texte était donc particulièrement attendu par nos concitoyens, par de nombreuses associations- cela a été dit -, et par les acteurs du secteur animalier. Le texte contient plusieurs dispositions ambitieuses, qui ont été conservées lors de la commission mixte paritaire : la création d'un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un animal de compagnie, l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie aux mineurs sans le consentement de leurs parents, la suppression de la vente des chats et des chiens en animalerie ou encore l'encadrement de la vente en ligne des animaux par l'instauration d'un label. Le renforcement des sanctions afin de lutter contre les actes de maltraitance et de zoophilie et limiter les abandons représente également une avancée indéniable.

à obtenir. Même si nous sommes tous favorables au bien-être animal, entre l'approche très pragmatique du Sénat et celle, volontariste, de l'Assemblée nationale, il paraissait complexe de trouver une issue commune. à force de concertation, de compromis, d'ajustements, en choisissant de minimiser les logiques partisanes au profit de l'intérêt de nos concitoyens et de la cause animale, nous y sommes parvenus.

le compromis trouvé prévoit l'interdiction des animaux sauvages dans un délai de sept ans après la promulgation de la loi, à condition que des solutions adaptées au bien-être des animaux existent. À défaut, un décret permettra aux cirques de conserver les espèces pour lesquelles des solutions acceptables n'auraient pas été trouvées. Dans les delphinariums, la détention de dauphins ne sera prohibée que d'ici à cinq ans. Les spectacles seront également interdits à terme. Néanmoins, la présence d'animaux reste possible dans les refuges, suivant des critères qui seront définis par arrêté, afin notamment de faire valoir leur dimension scientifique.

enfin la proposition commune sur l'encadrement strict des offres de cession en ligne des animaux de compagnie et la fin immédiate des élevages de visons pour leur fourrure. définitive, grâce à ce texte issu de la majorité présidentielle, nous apportons des mesures concrètes qui changeront le quotidien de nos animaux et amélioreront leurs conditions de vie. Il me semble utile d'ajouter qu'il est particulièrement constructif que le Sénat et l'Assemblée nationale puissent faire oeuvre commune sur des sujets aussi sensibles pour nos concitoyens,

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « le véritable test moral de l'humanité [ ...], ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci : les animaux Kundera a vu juste. Si nous ne luttons pas contre la maltraitance animale, personne ne le fera. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Il faut nous en féliciter, car ce texte est attendu par beaucoup de nos concitoyens. Il s'inscrit d'ailleurs dans une tendance de fond, qui s'est traduite par plusieurs initiatives législatives. La version sur laquelle le Parlement s'est accordé est un texte d'équilibre, qui prend en compte les réalités de notre pays. Près de la moitié de nos concitoyens possède un chat ou un chien. Nous ne pensons pas qu'un animal domestique soit un animal maltraité, comme le prétendent certains. L'histoire de l'humanité est intimement liée à celle des animaux. La relation entre l'humain et le chien remonte au moins à plusieurs dizaines de millénaires. Nous devons non pas renoncer à ces liens, mais mieux protéger les animaux contre les mauvais traitements.

Le texte prévoit à cet effet que les particuliers qui acquièrent un animal devront disposer d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Cette mesure peut paraître symbolique, mais elle permettra au moins de s'assurer que les fondamentaux sont connus. La proposition de loi renforce également l'encadrement de la vente d'animaux de compagnie. La vente sur internet sera désormais interdite, et c'est heureux : les animaux ne sont pas de simples marchandises. Les conditions de vente en animalerie sont également revues. Les animaux ne devront pas être visibles depuis la rue, afin de réduire les acquisitions impulsives. Nous nous interrogeons cependant, comme Mme la rapporteure, sur la pertinence d'une interdiction générale de la vente de chiens et de chats dans les animaleries.

La solution retenue est un entre-deux qui ne nous paraît pas satisfaisant. Ces professionnels méritent mieux. Ils peuvent être utiles à la lutte contre la maltraitance. Le texte leur confie d'ailleurs un rôle de promotion de l'adoption des animaux de refuges. Ces derniers sont en effet submergés par l'ampleur des abandons. Pour éviter l'échec que constitue l'euthanasie, nous devons trouver des solutions pour les 100 000 animaux abandonnés chaque année. À cet égard, nous saluons l'expérimentation permettant à l'État et aux collectivités de mieux se coordonner pour gérer les populations de chats errants. Ces populations sont en effet un sujet de préoccupation majeure pour de nombreuses communes, notamment dans le nord de la France, comme l'avait indiqué notre collègue Jean-Pierre Decool. Le texte prévoit aussi de lutter plus efficacement contre les importations illégales d'animaux. Ces trafics nuisent gravement à la condition animale, mais aussi à nos propres filières. Le montant de l'amende encourue est quadruplé, passant ainsi de 7 500 à 30 000 euros. Au-delà de la lutte contre l'abandon et ses conséquences, la proposition de loi renforce également les sanctions des actes de maltraitance. Certaines circonstances le justifient,

Je rappelle toutefois que la réponse pénale n'est certainement pas la panacée, que nos juridictions sont d'ores et déjà engorgées et que, malgré la hausse des crédits de la justice cette année, le nombre de magistrats n'a pas beaucoup augmenté depuis le siècle dernier.

il est important de rappeler ce matin que la protection des animaux n'est pas une préoccupation nouvelle. La France a posé dès 1850 le premier jalon d'une législation protectrice des droits des animaux domestiques en punissant d'une amende les mauvais traitements infligés publiquement. Cette législation s'est étoffée au fil des années jusqu'à reconnaître, en 2015, que les animaux étaient « des êtres vivants doués de sensibilité Aujourd'hui l'attente sociétale est grande pour aller plus loin dans la protection des animaux et moderniser en conséquence notre législation. Le texte proposé par l'Assemblée nationale, qui est le fruit de plusieurs initiatives parlementaires, n'est pas une loi structurante sur le bien-être animal. Toutefois, son périmètre réduit a permis à notre rapporteure, dont je veux saluer le travail, et à notre assemblée, de mener cette analyse de façon approfondie et dans des délais restreints. Le Sénat a veillé à amplifier les mesures qui lui semblaient aller dans le bon sens, à corriger les effets de bord de certaines propositions, à supprimer les dispositions qui n'étaient pas en phase avec la réalité des pratiques et, de façon générale, à maintenir une place pour les animaux dans notre société. En effet, la tentation est grande, pour certains, d'interdire à brève échéance toute détention d'animaux, voire même tout contact avec eux. Nous disons au contraire que la relation entre les animaux et les hommes fait partie intégrante de notre société. Loin de tout dogmatisme, le Sénat a souhaité valoriser dans ses propositions des solutions opérationnelles reposant sur des critères objectifs et scientifiques élaborés en lien avec les professionnels, les associations et et les vétérinaires, dans le but d'améliorer les conditions de vie des animaux. Je me réjouis que nombre de ces propositions aient été maintenues dans le texte final. J'en citerai quelques-unes, qui concernent les animaux domestiques. La reconnaissance du travail des associations sans refuge, d'abord : le texte issu de l'Assemblée nationale aurait entraîné la fin des activités des 3 200 associations sans refuge existantes, pourtant très actives et nécessaires sur le terrain. Sur l'initiative du Sénat, un statut juridique a été créé pour permettre à ces structures de poursuivre leur mission de prise en charge des animaux. la vente des animaux en animalerie. Une interdiction sèche de l'activité des animaleries n'était pas la solution aux problèmes soulevés par les députés : contrôles insuffisants, règles parfois inadaptées, achats impulsifs, nombreux abandons, défaut de formation des acquéreurs ... Elle aurait au contraire redirigé l'activité de vente vers des canaux certainement moins satisfaisants du point de vue du bien-être animal. pourquoi le Sénat a autorisé de nouveau la vente des animaux de compagnie dans les animaleries, à l'exception des chiens et des chats, encadré cette activité et encouragé les partenariats entre animaleries et associations de protection des animaux, dans le but de trouver une famille aux chiens et aux chats abandonnés. Je pense encore à l'encadrement de la vente des animaux domestiques en ligne. Face à ce qui est devenu la première animalerie de France, il est apparu indispensable au Sénat de fixer un cadre pour la vente des animaux domestiques en ligne, dans le double but de lutter contre les trafics et de s'assurer du bien-être des animaux proposés à la vente. Je pense enfin au renforcement des sanctions contre les maltraitances à l'encontre des animaux domestiques. Le Sénat a sensiblement amélioré le texte sur ce point, par exemple en créant des circonstances aggravantes en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté, en renforçant les plaintes en cas de vol d'un animal domestique lorsque ce vol est destiné à alimenter le commerce illégal, en réprimant plus fortement la zoopornographie, en créant un délit d'atteinte sexuelle sur animal domestique pour condamner la zoophilie. D'autres propositions tout aussi structurantes ont été maintenues. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera le texte issu de la CMP. Conformément

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Je voudrais vous dire qu'en la matière, le Gouvernement a tout de même fait une petite erreur de méthode. Une telle ambition méritait un projet de loi, « filtré » par le Conseil d'État et travaillé sérieusement en amont avec toutes les associations et les professionnels. Cela nous aurait évité de nous trouver face à un texte mal élaboré, sans et parfois contre les professionnels - je pense notamment à la façon dont les circassiens ont été particulièrement maltraités au début. Cette proposition de loi était mal préparée, parfois dogmatique pour être médiatique, et servir l'exposition de certains plutôt que le règne animal Pour ma part, je tiens à vous le dire, je n'ai jamais eu à examiner un texte dans de telles conditions. Je me réjouis néanmoins du travail qui a été effectué et du vote que nous venons d'obtenir, à la quasi-unanimité.

avec lesquels nous avons échangé sérieusement et de façon constructive, et les professionnels formidables que nous avons rencontrés, qui font sur le terrain un travail exceptionnel.

et cette proposition de loi a pu profondément les heurter et les blesser. Je veux leur dire le soutien total du Sénat. Nous porterons une attention particulière à la poursuite de leur activité et à l'avenir de leurs animaux. Mes chers

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (texte de la commission n° 84, rapport n° 83) et des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire

Ce texte, dont l'intitulé affiche l'ambition, est avant tout consacré à l'exercice des différentes professions judiciaires. En effet, si 53 % des Français ne font pas confiance à l'institution judiciaire, ils font majoritairement confiance à ses professionnels qui, malgré des conditions d'exercice souvent difficiles, portent cette institution

Si nous ne sommes toujours pas convaincus que ce texte composite permette à lui seul de restaurer la confiance, nous l'avons néanmoins examiné dans un esprit constructif, qui a permis de déboucher sur un accord en commission mixte paritaire Comme tout accord, celui-ci est imparfait, mais il reprend de nombreuses avancées adoptées par le Sénat, notamment la meilleure organisation de la discipline et de la déontologie des professions judiciaires, la force exécutoire pour les accords négociés entre avocats, l'enregistrement et la diffusion des audiences, ou la réforme des remises de peine et du travail pénitentiaire. De même, cet accord entérine des dispositions votées par le Sénat, qui correspondent aux standards que nous avions posés comme préalables, comme l'avertissement pénal probatoire, qui remplace le rappel à la loi. Concernant les cours criminelles départementales, nous avons obtenu le prolongement de l'expérimentation d'une année supplémentaire pour ne les généraliser qu'à partir du 1 janvier 2023, ce qui nous laissera le recul nécessaire. c'est ce texte de compromis, fruit de nombreux et intenses échanges avec nos collègues de l'Assemblée nationale, mais aussi avec M. le garde des sceaux, que nous vous soumettons aujourd'hui pour approbation. Certaines dispositions, notamment sur le secret professionnel des avocats, sont encore mal comprises. Mais je suis convaincue que les explications de mon collègue Philippe Bonnecarrère, qui n'a pas ménagé sa force de conviction et de pédagogie, éclaireront le sens des travaux du Sénat, et que la pratique lèvera les dernières résistances.

Vous avez pu constater que le Parlement, au terme du débat, écoutait les arguments, et l'accord que nous avons trouvé en CMP en a été pour vous la démonstration.

porte aussi sur les cours départementales criminelles et l'organisation déontologique des professions juridiques.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

... Ce second regard permet de prospérer ensemble. Ceux qui ont pu dire que nous étions en opposition sur certains sujets, et notamment sur le secret professionnel, se sont trompés. Sur ce point, je suis parti du secret de la défense ; les députés y ont ajouté le secret du conseil ; et le Sénat a rappelé, à juste titre, comme vous venez de le faire, monsieur le rapporteur, que le secret du conseil n'était pas absolu, qu'il n'était pas garanti par notre Constitution, contrairement au secret professionnel de la défense, car le conseil est une activité de services,

coconstruit le texte, et nous sommes parvenus à des solutions qui, me semble-t-il, sont de nature à restaurer la confiance. J'ai bien entendu qu'il ne suffit pas d'un texte, hélas ... Ce serait trop beau, ce serait la baguette magique que je ne partagerais avec personne ! Il ne suffit certes pas d'un texte pour rétablir la confiance, mais je voudrais revenir

du bon fonctionnement de la justice. Dans les dictatures, la justice n'est pas publique. Nous allons écarter les murs de l'audience. J'en viens à l'enquête préliminaire. Il n'est pas anormal que dans une grande démocratie comme la nôtre, on enserre l'enquête préliminaire, devenue parfois enquête éternelle, dans des délais. C'est une violation patente des droits de l'homme que de savoir qu'un homme peut être suspecté pendant deux, trois, quatre ans, parfois plus, sans savoir à quelle sauce il va être mangé, avec, parfois, quelques atteintes graves à sa présomption d'innocence dans la presse.

cas autrefois, il faudra désormais qu'une majorité de jurés se soient exprimés pour envisager une condamnation. En ce qui concerne des cours départementales, j'ai entendu ce qu'a dit le Sénat, lequel a souhaité que l'expérimentation se poursuive.

pourquoi pas ? Je n'ai pas du tout l'intention d'être caporaliste, et la voix des parlementaires m'importe infiniment. Pour que cette cour départementale, dont nous savons déjà qu'elle est efficace, soit mise en oeuvre et généralisée, nous allons donc attendre la fin de l'expérimentation. crimes en série, la réforme est extrêmement importante. Nous allons créer une juridiction nationale. Je pense à toutes les victimes qui n'ont pas connu n'ont pas connu ce qu'elles espéraient- l'interpellation, l'arrestation et le jugement des auteurs de crimes sériels -pour une raison absolument insupportable à nos yeux, qui

suppression du rappel à la loi, j'ai également entendu ce que disait le Sénat. Je proposais un an, vous en proposiez trois, nous avons retenu deux : quelle sagesse ! Ce rappel à la loi, plus personne n'en voulait. Il n'impressionnait plus que les honnêtes gens,

Permettre à une personne d'obtenir, sur une peine de dix ans, deux ans de réduction automatique sans aucun effort, c'est hérétique. C'est hérétique pour tous ceux qui travaillent ! Puis, le sens de l'effort n'est pas interdit : c'est bon pour le détenu, c'est bon pour ceux qui savent que le détenu sortira un jour,

Ils comprennent les avancées considérables qui ont été apportées tant au secret professionnel de la défense qu'au secret du conseil, dont nous parlerons dans quelques instants.

le projet de loi. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

le projet de loi. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.